Mais nous avions aussi considéré que l'habilitation demandée était trop large, puisqu'il s'agissait de transposer quatre directives et trois règlements européens

Ces textes européens procèdent à la refonte des critères relatifs aux biocarburants durables, aux performances énergétiques des bâtiments, à l'efficacité énergétique. Pourquoi n'en avons-nous pas débattu ?

Enfin, cet article de tarification a été introduit par voie d'amendement du Gouvernement lors des débats à l'Assemblée nationale. Ces dispositions

par un bioliquide renouvelable permettrait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation du fioul domestique. En effet, l'incorporation d'un bioliquide dans le fioul domestique entraîne une réduction de 50 % à 70 % des émissions de gaz à effet de serre Le développement de l'incorporation de ce bioliquide permettrait également de préserver le mode de chauffage des territoires les plus éloignés des grandes métropoles. Le fioul est aujourd'hui la troisième énergie de chauffage en France, équipant près de 4 millions de logements, dont 3,5 millions de résidences principales. Il est particulièrement utilisé dans des zones où les températures hivernales sont basses et où les réseaux de gaz n'existent pas. De plus, en soulignant la vulnérabilité de certains modes de fonctionnement de la mondialisation, la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 appelle notamment un renforcement de la souveraineté agricole française. Comme le souligne le plan Protéines végétales dévoilé le 1 décembre 2020 par le ministre de l'agriculture, la France est aujourd'hui dépendante des importations de protéines végétales. La création d'un débouché à la production d'ester de colza favoriserait donc l'indépendance protéinique de notre La filière industrielle d'estérification française est d'ores et déjà en capacité d'assurer l'approvisionnement nécessaire ; cette filière est en recherche de débouchés pour les huiles résultant de la trituration.

présent amendement a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat. ordonnance prévoit, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, l'obligation d'installer des systèmes d'automatisation et de contrôle dans les bâtiments tertiaires les plus consommateurs, ainsi que des dispositifs de régulation de la température par pièce dans tous les bâtiments résidentiels et tertiaires en cas d'installation ou de modification d'un générateur de chaleur. L'ordonnance prévoit également d'améliorer l'information individuelle des ménages sur leur consommation d'énergie lorsqu'ils occupent un logement dont le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire sont collectifs, des ménages abonnés à un réseau de chaleur. Enfin, elle étend aux systèmes de chauffage, dont les pompes à chaleur et les chaudières biomasse, les obligations d'inspection et d'entretien déjà en vigueur pour les chaudières au gaz et au fioul.

unique en matière de stratégie énergétique pour les territoires des zones non interconnectées, dont font notamment partie les territoires ultramarins. Elle précise les objectifs de politique énergétique, identifie les enjeux et les risques dans ce domaine et oriente les travaux des acteurs publics. La PPE couvre deux périodes successives de cinq ans qui permettent de piloter le système énergétique de ces territoires, en tenant compte de l'évolution des techniques, du contexte économique et des enjeux sociaux et environnementaux locaux. Elle contient par ailleurs des outils de pilotage financier. Cet amendement vise à instituer une évaluation de l'application des des objectifs et des coûts financiers de la PPE à mi-parcours, soit tous les trente mois.

la PPE définit un ensemble d'indicateurs qui répondent au même objectif et qui sont suivis régulièrement. Enfin, l'impact financier des dispositifs de péréquation et de soutien aux énergies renouvelables fait l'objet d'une présentation au Parlement

Cet amendement vise à porter la part maximale de prise en charge par le tarif de réseau à 60 % dans le cas des installations de production d'électricité renouvelable de petite taille. Le Gouvernement s'assurera, lors de l'adoption de l'arrêté fixant les nouveaux taux de réfaction, que l'économie générale des dispositifs de soutien tarifaire n'est pas significativement modifiée. Par ailleurs, l'évolution des besoins liés à la consommation d'électricité, tels que l'installation d'une pompe à chaleur, peut conduire à des travaux substantiels, notamment de remplacement ou d'adaptation de certains ouvrages sur le réseau public d'électricité. Le demandeur du raccordement doit alors payer une contribution au coût de ces travaux, qui peut s'avérer dissuasive pour l'installation des dispositifs. Cet amendement a donc pour objet de lever ces obstacles, pour que les citoyens puissent s'approprier le développement des énergies renouvelables. Cette mesure

Le niveau de prise en charge sera précisé par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE. Il pourra, le cas échéant, être inférieur à 100 %. De plus, la liste des opérations pouvant faire l'objet d'une telle prise en charge sera définie par décret, également pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

souvent très difficile, parce qu'elle doit passer par différentes étapes administratives, notamment des enquêtes publiques, d'une part, et des autorisations d'urbanisme, d'autre part.

en effet, insister sur la nécessité de développer une méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité, à l'échelle de son patrimoine et de ses compétences, qui intègre la forme de la fourniture

la loi Royal, sur la nécessité pour l'État de fournir aux collectivités des méthodologies simplifiées sur leur bilan de gaz à effet de serre- non pas celui qui est lié au patrimoine et aux compétences, mais plutôt le bilan Scope 2 sur l'ensemble des émissions du territoire. À ma connaissance, on attend encore ... Quel est l'avis de la commission économiques ? L'indication du mix énergétique dans les plans de transition n'est pas souhaitable. En effet, ceux-ci prévoient déjà que les collectivités territoriales ou leurs groupements précisent les objectifs, moyens et actions.

est ainsi libellé : La parole est à M. Daniel Salmon. Aujourd'hui, la majorité des bâtiments existants ne sont pas solarisables, parce que les contraintes techniques qui auraient permis leur solarisation n'ont pas été envisagées au moment de la construction. Pour permettre l'indispensable déploiement de l'énergie solaire, il est essentiel d'éviter ce problème pour les futurs bâtiments qui vont être construits. Il faut donc faire en sorte que toutes les futures constructions neuves soient solarisables, même si l'installation ne se fait pas immédiatement. Pour ce faire, il faut, lors de la construction, tenir compte des charges supplémentaires apportées à la structure par une éventuelle installation solaire. On pourra également envisager l'intégration de l'installation en harmonie avec les autres équipements présents sur la toiture. S'il existe un léger surcoût à la construction d'un bâtiment solarisable par rapport à un bâtiment qui ne l'est pas, on estime que celui-ci représente entre 1 % et 3 % du budget alloué à la construction du bâtiment.

pour déterminer les conditions techniques d'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques. Il s'agira de préciser que la rénovation doit prévoit d'accueillir ces panneaux. Par ailleurs, la rédaction proposée écarte une grande partie des modes constructifs des bâtiments tertiaires, en visant uniquement les constructions de type charpente. C'est pourquoi je maintiens l'avis défavorable

est ainsi libellé : La parole est à M. Jean-François Longeot. Faute de ressources foncières suffisantes, le parc solaire français ne progresse que d'un gigawatt par an, ce qui est largement inférieur aux ambitions fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie, Or, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, les zones naturelles, agricoles et forestières, ne peuvent plus en principe accueillir de centrales photovoltaïques au sol. L'interdiction est générale et sans exception. Seules les zones délaissées et artificialisées sont autorisées à accueillir des centrales photovoltaïques. Dans ces conditions, l'objectif de 20,6 gigawatts de puissance installée en 2023, avec une cible de 35,6 gigawatts à 44,5 gigawatts en 2028, semble hors d'atteinte. Or le déploiement de petites centrales photovoltaïques à faible impact environnemental, raccordées au réseau à basse tension, permettrait de mailler le territoire en milieu diffus Ce déploiement serait d'autant plus facile que des installations de type ou ombrières constituent une réponse efficace à la pression foncière, permettent de tenir l'ambition de réduction de l'artificialisation des sols, en réduisant l'emprise au sol, et favorisent l'agrivoltaïsme, qui concilie la préservation des terres agricoles et la mise à profit de surfaces foncières pour le développement des énergies renouvelables. Le présent amendement vise à prévoir l'installation de centrales solaires dont l'emprise au sol est minime, dont le déploiement ne se fait aucunement au détriment d'une autre activité, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Quel

suite à l'expérimentation proposée, qui vise à autoriser l'implantation d'installations photovoltaïques dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. D'une part, les dérogations seraient très larges. D'autre part, les zones de revitalisation rurale ou celles qui ont 80 % de surfaces agricoles ne sont pas forcément les mieux adaptées à la réalisation des projets.

objet de renforcer l'impact des achats publics sur la transition énergétique, en proposant aux acheteurs publics des critères concrets à forte plus-value environnementale et sociétale. C'est un sujet dont nous avons déjà eu l'occasion de débattre. Quel est l'avis de la commission

le développement des communautés d'énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.

a fait référence à la loi Énergie-climat du 8 novembre 2019, qui associe tous les types d'énergies renouvelables.

madame la ministre,

Par ailleurs, rien ne justifie que les projets d'implantation d'éoliennes spécifiquement portés par les communautés d'énergie renouvelable bénéficient d'un traitement fiscal préférentiel. L'avis de la commission

la transition énergétique est régulièrement évoquée, nous constatons que sa traduction sous forme de dispositions réglementaires concrètes n'est pas encore au rendez-vous. La décentralisation de la production d'énergies renouvelables adaptées aux ressources locales offre la possibilité à des acteurs locaux de devenir producteurs d'énergie et acteurs de la transition énergétique.

pour favoriser l'émergence des projets gérés par ces acteurs territoriaux et faire de l'implication citoyenne dans les énergies renouvelables la clé de la réussite en matière de transition énergétique. Sur le plan opérationnel, il s'agit de travailler à la bonne articulation entre les différents échelons de planification, pour mettre en cohérence les objectifs et les dispositifs de soutien à ces projets. Mes chers collègues, je suis persuadé qu'il existe près de chez vous un certain nombre de projets locaux de production d'énergie renouvelable,

Conformément à la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, la part des énergies renouvelables doit représenter 33 % de la consommation finale en France en 2030, objectif qui ne sera pas atteint si le développement des énergies renouvelables se poursuit au rythme actuel, comme M. Longeot l'a rappelé tout à l'heure.

et ce pour au moins 50 % de leur surface totale. Il tend également à inciter plus fortement à l'installation, au choix, de toits végétalisés ou d'un dispositif photovoltaïque sur les constructions à venir. Le couplage des deux solutions peut également être envisagé, en tenant compte de la plus forte capacité de rafraîchissement des dispositifs végétaux, d'une part,

Je partage votre objectif, mon cher collègue, à savoir renforcer les dispositions environnementales relatives à certains parcs de stationnement. Ces mesures sont cohérentes avec le travail effectué et les modifications adoptées à l'article 24, en matière de périmètre comme pour les actions qui doivent être effectuées. J'émets toutefois une réserve sur les obligations proposées, dans la mesure où celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une évaluation, tant de leur impact économique que de leur impact environnemental. Mon interrogation porte notamment sur l'obligation de couvrir la totalité

Pour d'évidentes raisons géographiques, ces sites sont particulièrement nombreux dans les départements et régions d'outre-mer, les DROM, où les communes soumises à la loi Littoral peuvent s'avancer loin dans les terres. Le présent amendement vise à harmoniser le régime applicable en métropole et dans les DROM, en modifiant le code de l'urbanisme pour autoriser l'implantation de centrales solaires au sol

Cet amendement vise à étendre le dispositif introduit en commission à l'article 24 , afin d'en prévoir l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Par cohérence avec la position qui était la mienne lors de l'examen du texte en commission, je m'en remets à la sagesse

Faire coopérer les associations environnementales, les entreprises, les syndicats, les pouvoirs publics pour une transition socialement acceptable et économiquement tenable est indispensable. Je constate, en voisin, combien l'exécutif écologiste du Bade-Wurtemberg parvient à travailler de façon étroite avec les constructeurs.

fondée sur une trajectoire et un budget carbone sérieux, accompagnés de compensations réelles. Nous souhaitons un basculement net vers le rail et la réduction des avantages fiscaux et tarifaires contre-productifs dont

qui pourrait nous faire économiser 1,4 million de tonnes de CO2. Reste encore à améliorer le forfait mobilité durable et à encourager les stationnements sécurisés. Enfin, il ne serait pas raisonnable de décaler de cinq ans la mise en place des ZFE.

commission. S'agissant de l'article 25, nous faisons face collectivement à une véritable révolution, en tout cas à une transition très rapide dans le champ de la mobilité électrique.

socialement soutenable, en tout cas acceptable. C'est dans cet état d'esprit global que nous nous trouvons aujourd'hui ; plus généralement, c'est l'état d'esprit qui nous anime pour examiner ce titre III relatif aux mobilités.

Le présent amendement vise à prendre en compte l'analyse de cycle de vie des énergies utilisées. En effet, l'article 25 modifie l'article 73 de la loi lequel précise que l'objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d'ici à 2050 s'entend sur « le cycle carbone de l'énergie utilisée Le seuil de CO2 auquel fait référence l'article 25 s'appuie néanmoins sur la mesure des émissions de CO2 au pot d'échappement utilisée dans la réglementation européenne, qui, à elle seule, est insuffisante pour quantifier l'impact des émissions d'une voiture sur le climat.

les carburants à essence consommés contiennent de plus en plus de bioéthanol renouvelable issu des plantes ; cette particularité, bonne pour l'environnement, doit être prise en compte dans l'évaluation des émissions d'un véhicule. En effet, la combustion du bioéthanol renvoie à l'atmosphère le CO2 absorbé par les plantes pour leur croissance, et ce cercle vertueux n'augmente pas l'effet de serre.

la commercialisation des voitures neuves émettant plus de 123 grammes de CO2 par kilomètre, selon la norme WLTP. La commission des affaires économiques a adopté, à juste titre, un amendement tendant à préciser que le soutien de l'État comprend notamment le recours aux biocarburants. Il convient donc de ne pas freiner certaines filières, telles que le superéthanol E85. Or les mesures d'émissions retenues par la réglementation européenne ne permettent pas, à elles seules, de quantifier les émissions de gaz à effet de serre des voitures. L'analyse du cycle du carbone de l'énergie utilisée doit être prise en compte en ce qui concerne le superéthanol E85, dont la combustion renvoie dans l'atmosphère le dioxyde de carbone. Le présent amendement vise à prendre en compte cette particularité en prévoyant l'application d'une réduction de 40 % sur les niveaux d'émissions de dioxyde de carbone pour les voitures particulières neuves dont la source d'énergie comprend le superéthanol E85. Le recours à ce biocarburant constitue un atout intéressant pour la transition écologique du parc automobile, ainsi que pour le porte-monnaie de nos concitoyens, le prix à la pompe de ce carburant étant actuellement de 0,66 euro le litre.

aval, considérablement affectées par cette transition industrielle. En fixant dès à présent l'échéance à 2030, nous donnerons de la visibilité aux constructeurs, nous améliorerons les conditions d'anticipation et d'accompagnement des impacts sur l'emploi, la transformation des métiers et la gestion des compétences.

Les carburants à essences consommés contenant du bioéthanol renouvelable issu de plantes contribuent à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Cette particularité doit être prise en compte dans l'évaluation des émissions d'un véhicule.

à cette même date la fin de la vente de poids lourds, d'autobus et d'autocars neufs utilisant majoritairement des énergies fossiles. Pour accompagner ces évolutions, il est prévu un soutien à l'acquisition de véhicules propres.

lorsqu'ils ne favorisent pas une concurrence avec les cultures vivrières, contribuent eux aussi à des émissions de gaz à effet de serre ; ils n'offrent donc pas toujours un bon bilan carbone. En outre, leur production même peut consommer beaucoup d'énergie et dégrader leur bilan énergétique. Pour ces raisons, nous estimons nécessaire de préciser

Si l'échéance de 2030 fixée à l'article 25 permet aux constructeurs et aux industriels de visualiser une trajectoire claire, qui dynamisera le marché des véhicules à faibles émissions et permettra d'anticiper l'objectif fixé par l'Union européenne à 2040, il n'en est pas de même pour les professionnels de la réparation. Ces derniers devront s'adapter très rapidement, non seulement à un parc de véhicules thermiques vieillissant et à la possibilité de transformer les véhicules, mais aussi à l'arrivée de nouvelles énergies et, avec elles, de nouvelles technologies. Or ces véhicules, une fois sur le marché, devront être entretenus et réparés de manière optimale, d'après-vente, afin de conserver leur performance environnementale et de préserver la sécurité. Dès lors, la digitalisation et la modernisation des entreprises, nécessaires

: de nombreux véhicules peuvent fonctionner avec des biocarburants, mais également avec des carburants conventionnels ou avec des essences ayant une faible teneur en biocarburant au regard de nos objectifs de transition. Il n'est donc pas garanti qu'une telle dérogation bénéficie aux biocarburants.

Les enjeux de disponibilité de véhicules appropriés aux activités de montagne ou aux activités agricoles ne sont pas de la même ampleur que pour les véhicules lourds.

de l'amendement n° 94 rectifié, monsieur Demilly, il me semble important de reconnaître le caractère vertueux des biocarburants, qui ressort lorsque l'analyse de leurs émissions prend en compte leur cycle de vie.

d'expliciter que le recours aux biocarburants doit être un levier de décarbonation. Veillons à ce que toute précision allant dans ce sens ne soit pas prise

nos concitoyens pour que le report modal de leurs mobilités ne soit pas bloqué par des coûts insupportables et des inégalités de moyens rendant cette transition hors de portée des ménages populaires. le présent texte évoque ces aides au report vers des solutions de mobilités vertueuses : cet amendement tend à clarifier les modalités et le périmètre d'application des aides par voie de décret, au plus tard dans les six mois. Il s'agit de définir un cadre incitatif et rassurant permettant à nos concitoyens de choisir leurs nouvelles solutions propres de mobilité- vélo, vélo à assistance électrique, transports en commun, autopartage ou covoiturage

dernières incluent-elles les vélos-cargos, les vélos pliants, les services vélo, les abonnements aux transports en commun, les services d'autopartage ou encore de covoiturage

Le montant de ces aides est un enjeu crucial : il s'agit de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.

La logique serait ainsi celle d'un budget mobilité, avec un montant crédité sur un titre mobilité et des services de mobilité sélectionnés disponibles pendant plusieurs années- en

n° 1024 rectifié. L'Assemblée nationale a élargi le soutien à l'acquisition de véhicules propres, en particulier de vélos à assistance électrique, à la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique ou encore à l'installation d'équipements techniques destinés à améliorer la sécurité.

cet amendement, est de développer la filière de l'électromobilité, afin de suivre une trajectoire de décarbonation des véhicules terrestres. Ainsi, nous proposons d'ouvrir les données liées à la gestion de l'énergie des véhicules aux professionnels de la recharge pour voitures électriques, sous réserve du consentement des utilisateurs. L'ouverture de ces données permettra le développement de solutions et de services pour l'optimisation de l'énergie. Elle contribuera ainsi à la décarbonation du secteur des transports au cours des années à venir

ordonnance désormais publiée ne traduit pas fidèlement l'intention du législateur. L'extension de l'accès aux données aux services de l'automobile ou de développement de services innovants est la bienvenue : c'est la raison pour laquelle nous sommes favorables

Il s'agit notamment d'accompagner les artisans dans une démarche de verdissement de leurs véhicules. Si nous sommes favorables à cette disposition, nous jugeons nécessaire que ces aides soient ciblées au profit des ménages et artisans aux revenus modestes. L'enveloppe des aides et primes à la conversion n'étant pas extensible, elle doit être réservée en priorité aux ménages modestes : le « quoi qu'il en coûte » ne durera pas éternellement.

témoigne le prêt à taux zéro sous conditions de ressources pour l'achat de véhicules propres. Toutefois, si votre amendement était adopté, tout dispositif de report modal, qu'il concerne les motorisations décarbonées actives ou le report vers les transports en commun, serait réservé aux ménages ne dépassant pas un plafond de ressources. Il ne me semble pas nécessaire

Aussi, uniformiser l'action de l'État sur l'ensemble du territoire sans prendre en compte les différences entre le monde rural et le monde urbain est une grave erreur. Ce choix conduira inévitablement à des situations ubuesques dans nos territoires ruraux : les dispositions de ce projet de loi ne doivent pas être pensées selon le prisme métropolitain.

Cet article amplifie les dispositifs d'accompagnement des ménages dans les zones à faibles émissions mobilité, les ZFE-m, en complément des aides déjà prévues. Le périmètre de ces aides mérite d'être précisé : inclut-il les vélos-cargos, les vélos pliants, les services vélos, les abonnements aux transports en commun, les services d'autopartage et de covoiturage ?

plusieurs années-

Alors que la transition environnementale a un coût, l'État doit accompagner davantage les Français. Force est de constater, et vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, que s'il existe des dispositifs, ceux-ci ne sont pas suffisants. L'article 26 A, rédigé de concert avec la commission des finances,

Il n'en demeure pas moins que l'écart de prix à l'acquisition entre des véhicules propres et des véhicules thermiques reste très important. Un prêt à taux zéro permettra d'accompagner les ménages dans le renouvellement de leur véhicule. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement du Gouvernement.

un échelonnement des aides pour accompagner les ménages plus ou moins modestes. Il faut absolument que l'on ait une lisibilité, une visibilité sur ces questions. Aujourd'hui, l'industrie automobile et les industriels sont prêts. Ils vont

et à modifier sensiblement l'équilibre voté en commission. La restriction à des véhicules de moins de 1,3 tonne nous paraît contre-productive, car elle frapperait en premier lieu les familles nombreuses,

y compris dans les métropoles les plus densément peuplées. Je pense notamment à la question des ZFE, que nous aborderons plus tard. Par ailleurs, ces aides sont complétées en fonction

Aujourd'hui, les personnes utilisant une voiture privée pour se rendre sur leur lieu de travail bénéficient d'une indemnité kilométrique. Cet avantage fiscal, qui permet de déduire de l'impôt sur le revenu les frais de carburant dédiés aux déplacements professionnels, représente un montant d'environ 2 milliards d'euros

la voiture pour se déplacer. Actuellement, cette indemnité kilométrique dépend de deux facteurs : la distance parcourue et la puissance du moteur du véhicule. Autrement dit, le barème actuel des indemnités kilométriques favorise les véhicules puissants, donc plus émetteurs. Cette disposition est en contradiction avec les objectifs environnementaux. Elle constitue en outre un enjeu important pour les finances publiques, puisque les frais kilométriques représentent, je l'ai dit, près de 2 milliards d'euros chaque année dans le budget de l'État.

Nous proposons donc d'indexer l'indemnité kilométrique sur les émissions de CO2 de la voiture. Plus la voiture émet, moins l'indemnité sera élevée. Monsieur Moga, je comprends la philosophie de votre amendement et sa pertinence. Le forfait kilométrique est un outil servant au remboursement des frais d'utilisation d'un véhicule pour des raisons professionnelles. Il est donc indexé sur la consommation énergétique du véhicule et, de fait, sur sa puissance fiscale. La suppression de la prise en compte des chevaux fiscaux ne paraît pas opportune, dans la mesure où elle est nécessaire au calcul fidèle de la consommation du véhicule et au remboursement des frais de déplacement réels. De plus, une telle suppression aurait des conséquences importantes sur les exonérations fiscales relatives aux frais de déplacement. Je vous demande donc de bien vouloir retirer

est française. Pour rouler avec du superéthanol, il convient d'intégrer un boîtier bioéthanol, dont l'installation coûte entre 700 euros et 1 200 euros.

À cet égard, nous avons précisé en commission que les aides à la transition énergétique s'appliquent notamment à la transformation des véhicules et au développement des biocarburants. Le dispositif de conversion des véhicules à motorisation essence

que pour un vélo ou un vélo-cargo utilisé à des fins professionnelles. Une telle réduction inciterait au report modal, particulièrement pour la logistique urbaine et les derniers kilomètres de livraison. Elle faciliterait enfin le développement de la filière du vélo. Quel est l'avis de la commission ? Le secteur

La transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l'environnement passe par l'achat de véhicules plus propres. C'est pour cette raison qu'une prime à la conversion est versée aux citoyens lors de l'achat d'un véhicule moins polluant

C'est un gaspillage de ressources important. La destruction de ces véhicules ne participe pas à une lutte efficace contre le dérèglement climatique. En effet, la construction de nouveaux véhicules nécessite l'utilisation de ressources naturelles, de minerais, dont l'extraction génère l'émission d'importantes quantités de gaz à effet de serre.

à mettre à disposition des régions les véhicules destinés à la casse sous réserve qu'ils n'émettent pas une quantité de CO2 supérieure à un seuil qui serait défini après avis de l'Ademe. L'octroi de la prime à la conversion ne serait donc plus systématiquement conditionné à la destruction automatique du véhicule ancien. Les régions, qui ont déjà la faculté de mettre en place des services de location sociale de véhicules, pourront ainsi

je vous remercie

proposés concernent le tarif unitaire, déterminé en fonction d'un barème progressif, la diminution du seuil minimal de la taxe à 1,3 tonne et l'élargissement du champ d'application de la taxe aux véhicules électriques et hybrides rechargeables selon un barème et un seuil minimal spécifiques.

2,6 % des ventes de véhicules. Cet amendement vise donc à augmenter le malus poids, afin d'enrayer la dérive du marché automobile à l'oeuvre

pour entretenir la frénésie de consommation de grosses voitures. Les constructeurs automobiles de l'avenir seront ceux qui sauront opérer à temps la transition vers des modèles sobres et légers- ce sera la clé de la mobilité du XXI siècle mettre en place un malus poids à la hauteur des enjeux. Je pense que le meilleur service à rendre à notre industrie automobile est de la placer à la pointe de la transition.

tel renforcement de la taxe paraît en contradiction avec le plan de soutien à la filière automobile. Alors que les différents malus appliqués à l'automobile sont déjà importants,

d'aérodynamisme, de frottement minimal avec l'air et, par voie de conséquence, d'efficience en matière de consommation de carburant. Toutefois, si ce coefficient occupe une importance capitale dans le domaine de l'automobile, l'intérêt des constructeurs, qui communiquent moins sur cette donnée, décroît depuis plusieurs décennies.

L'installation systématique de services vélo dans les parcs de rabattement s'impose pour conforter le bond en avant du vélo, pour compléter le déploiement en cours de réseaux express vélo à l'échelle des agglomérations- cela se pratique à Paris, Strasbourg, Lyon ou encore

dans les parcs de rabattement situés en entrée d'agglomération ou à leurs abords. Le déploiement de ces stationnements vélo, associé à une politique de limitation du stationnement et de l'accès motorisé en centre-ville, doit permettre aux usagers du parc relais de réaliser les derniers kilomètres de leurs trajets quotidiens à vélo et contribuer à limiter la place de la voiture en ville. Notre proposition répond aux objectifs de la Convention citoyenne pour le climat

l'intermodalité, en incluant le vélo. S'il est nécessaire de promouvoir le rapport modal de la voiture vers les transports collectifs en entrée de ville les parcs de rabattement, il est également possible de favoriser une chaîne de mobilité

Le cadre réglementaire et législatif laisse des marges tout à fait importantes pour définir ce qu'est un plan de mobilité. Il y a déjà des objectifs sur le vélo et des sous-objectifs sur sa sécurisation. C'est

transports du quotidien dans notre pays. Cette transition suppose d'encourager très fortement le développement des parcs de rabattement ou parkings relais près des gares ou aux entrées de ville. C'est l'objectif de l'article 26. En revanche, dans des zones urbaines comme la métropole parisienne, où le foncier est rare, encourager les citoyens à privilégier les transports en commun plutôt que leur véhicule thermique suppose surtout de développer des stationnements sécurisés pour les vélos et autres engins de déplacement personnel. Aujourd'hui, les plans de mobilité ne sont pas censés être prescripteurs sur le développement de ces espaces. Cet amendement tend donc à renforcer la planification de la construction de stationnements sécurisés pour les vélos en prévoyant que les plans de mobilités des AOM définissent le nombre de places de stationnements de ces parcs vélos, exactement comme l'article 26 le prévoit pour les parkings relais. Par ailleurs, cet amendement vise à préciser que les plans de mobilité déjà approuvés par les AOM doivent obligatoirement être révisés d'ici à 2023 pour mettre en oeuvre les ambitions de l'article 26 sur le renforcement des parkings relais et des parcs vélos sécurisés.

de nature à renforcer la qualité des plans de mobilité. Par ailleurs, je ne suis pas favorable à une obligation de révision partielle de tous les plans de mobilité par toutes les AOM pour introduire une telle précision. Ce serait sans doute un peu trop lourd, même si je comprends le sens de cet amendement. En

Les enquêtes, qui ont lieu seulement tous les dix ans, procèdent par échantillons, avec des marges d'erreur assez importantes, sans prendre en compte les déplacements ponctuels, notamment les trajets à but touristique. Nous avons besoin d'une étude rigoureuse des déplacements par véhicule individuel pour permettre aux autorités organisatrices de la mobilité de comprendre les besoins des usagers et de rechercher toutes les alternatives crédibles à la voiture, dans l'objectif de faire évoluer les comportements de chacun. Cet amendement entend donc rendre accessibles aux AOM les données d'usage détenues par les assistants de déplacement numériques comme les calculateurs d'itinéraires routiers multimodaux de type GPS. La dynamique de ces informations permettra de mieux caractériser les besoins de déplacement et d'évaluer de façon réactive et précise l'impact des politiques publiques de mobilité.

Le plan de mobilité employeur prévu dans le code des transports vise à optimiser l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Je rappelle que le PDM évalue l'offre de transports existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels,

Le programme d'actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle- utilisation des transports en commun, covoiturage, autopartage, marche ou usage du vélo -, mais aussi

Il me paraît peu opportun d'étendre le périmètre de ces plans à d'autres entreprises, alors que nous ne disposons pas encore d'un recul suffisant sur leur efficacité et leur pertinence. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable monsieur le ministre,

aident à mettre en place les plans de mobilité employeur en accompagnant les entreprises. Il prévoit des sanctions en cas de non-transmission du plan de mobilité employeur par l'entreprise à l'autorité organisatrice de la mobilité correspondante dans un délai d'un an après la communication du plan de mobilité de l'AOM à l'entreprise. Cette concertation entre AOM et entreprises doit permettre d'aboutir à des plans de mobilité employeur compatibles

possibilité pour des TPE-PME de se raccrocher au plan de mobilité d'une entreprise plus grande située à proximité. L'objectif est de construire une cohérence de la mobilité à l'échelle d'un territoire, en mettant en place des solutions robustes et propres

La crise sanitaire a incité de nombreux employeurs à réfléchir aux modes de déplacement de leurs employés, notamment en promouvant les mobilités douces. Cette prise de conscience peut être favorisée par l'élaboration d'un plan de mobilité. Pour autant, les petites entreprises ne sont pas soumises à l'obligation d'élaborer un tel plan. D'ailleurs, les employeurs à qui elle incombe ne la respectent pas systématiquement, ce qui n'est guère étonnant étant donné l'absence de sanctions prévues en cas de non-respect de l'article L. 1214-8-2 du code des transports. Inspiré par une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, cet amendement vise à inciter les administrations et les entreprises à mieux organiser les mobilités de leurs salariés ou agents dans une optique de réduction du CO2.

les dispositions concernées sont récentes, puisqu'elles sont entrées en vigueur le 1 janvier 2020 seulement. Il faut peut-être se donner le temps de mettre en place les plans de mobilité employeur et de procéder à un retour d'expérience sur la durée.

Les organisations syndicales comme patronales se sont exprimées défavorablement sur l'idée de rendre obligatoire le plan de mobilité employeur, ce qui ramènerait à la situation antérieure. Les partenaires sociaux ne souhaitent pas

Cette solution constituerait un trait d'union entre la ligne de bus et le covoiturage classique. Les conducteurs seraient incités à emprunter cette ligne préférentielle, qui disposerait de points d'arrêt fixes et sécurisés pour les covoiturés.

matière. Les autorités organisatrices de la mobilité sont aujourd'hui compétentes pour organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules particuliers ou contribuer au développement de ces usages.

émettra un avis défavorable.